en permettant aux agents de sécurité des transports d’intervenir aux abords immédiats de la gare, alors même qu’aucune infraction

d’actes terroristes aux abords immédiats des gares, y compris en l’absence d’autorisation préfectorale. Il ne fait guère de doute qu’une telle faculté constitue une prérogative de police administrative générale et serait regardée comme telle par le Conseil Ainsi, une telle mesure est très clairement contraire à l’interdiction de la délégation à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la force publique. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

que, « dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche ». Le Gouvernement considère donc que cet amendement est satisfait et en demande le rejet.

la fois troubler l’ordre public et avoir un comportement compromettant la sécurité des personnes ou la régularité de la circulation. Le présent amendement vise à rendre ces conditions alternatives. Je n’y suis pas opposée

de déplacement, alors même que le renforcement de leur attractivité, dans une logique de report modal, constitue l’un des objectifs cardinaux de la proposition de loi.

est une fausse bonne idée.

En deuxième lieu, ces amendements tendraient à créer une différence de traitement entre agents de la Suge en fonction de la filiale à laquelle ils sont rattachés, sans que cette différence soit justifiée par des différences objectives de situation. En dernier lieu, cette évolution reviendrait à confier à certains agents de la Suge, qui – je le rappelle – sont des agents de sécurité privée, les mêmes prérogatives que les forces de sécurité intérieure sur la voie publique, ce qui est à l’évidence en rupture avec la cohérence du continuum de sécurité dans les transports.

du Gouvernement ? Dans une décision du 31 mars 2023, le Conseil constitutionnel a rappelé que, pour procéder à des constatations donnant lieu à procès verbal, les agents contractuels de droit privé devaient être commissionnés et assermentés. Les dispositions proposées dans ces amendements seraient donc contraires à l’article 66 de la Constitution,

à cet article, qui permet le libre accès des agents de la police municipale aux espaces et matériels roulants des transports de voyageurs, aux espaces de transport et aux trains en circulation. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 20 mai 2021 sur la loi Sécurité globale, a émis plusieurs réserves d’interprétation et une censure concernant des mesures appliquant le continuum de sécurité, notamment en ce qui concerne les prérogatives de la police municipale. « résulte de l’article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire. Cette exigence ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d’enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents

pour être habilités à exercer leurs missions de police judiciaire, suivre une formation et satisfaire à un examen technique selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, il n’est pas prévu qu’ils présentent des garanties équivalentes à celles qui sont exigées pour avoir la qualité d’officier de police judiciaire

La commission considère, à l’inverse de leurs auteurs, que des synergies et des complémentarités doivent être trouvées entre les différents acteurs du continuum de sécurité. Il appartient aux acteurs publics de veiller collectivement à ce que les contrevenants ne puissent jouer avec des frontières administratives pour semer les agents de la police municipale. En la matière, la commission a néanmoins veillé à réaffirmer l’autorité du maire sur l’action de la police municipale.

? J’ai envie de réconcilier les amoureux… Mon avis sera favorable ! En effet, l’article L. 511 1 du code de sécurité intérieure permet d’ores et déjà aux policiers municipaux d’intervenir, sous l’autorité sous l’autorité du maire, dans les espaces de transport, dans le cadre de la signature d’une convention locale de sûreté dans les transports collectifs. À Dunkerque, j’en ai été le témoin privilégié, dernièrement, quand j’ai pris le train : c’est bien la police municipale

Dois je vous rappeler qu’il était question, dans cette décision, de l’extension des prérogatives de police judiciaire aux policiers municipaux ? Or il n’est nullement question, ici, de leur confier des prérogatives de police judiciaire ; il s’agit plutôt de leur accorder des prérogatives de sécurisation des véhicules de transport.

de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers ». Ce dispositif est donc mis en œuvre à compétences constantes. L’audition des responsables d’IDFM que j’ai conduite a d’ailleurs mis en évidence, à ce titre, le renforcement en cours des services chargés de la sûreté au sein de cet établissement, dans la perspective

pour faciliter la coordination de l’action des services internes de sécurité des opérateurs autres que la RATP avec celle des forces de sécurité intérieure. La préfecture de police souscrit pleinement à cette initiative, qui est attendue.

la tarification des prestations réalisées « en monopole » par le GPSR serait déterminée dans le cadre de la convention bilatérale entre IDFM et la RATP, sans référence à ce document. Je ne crois vraiment pas que ce texte soit le véhicule adéquat pour ce type de mesures, qui relèvent, au fond, des relations financières entre IDFM et la RATP.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

entre autres. Enfin, l’expérimentation a démontré que dans certains cas, la caméra piéton pouvait être activée à la demande de l’usager contrôlé. Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission est donc défavorable.

des images captées par la RATP et la SNCF aux centres de supervision urbains de la police et de la gendarmerie nationale. L’amendement n° 17 rectifié est, en pratique, pleinement satisfait en région Île de France, où ce rôle est joué par le CCOS

L’auteur de l’amendement semble en avoir conscience, puisque son dispositif prévoit bien que cette transmission soit mise en œuvre « lorsque cela est raisonnablement réalisable

et la mise en relation avec d’autres traitements. Cependant, le traitement algorithmique est une technologie qui prévoit un traitement automatisé d’informations par l’intelligence artificielle, avec ses biais et ses risques sociétaux. Nous atteignons ici la limite

Soyons raisonnables et mesurés. Ces nouvelles solutions techniques seront utilisées dans le pays lors des jeux Olympiques. Attendons de connaître leur efficacité réelle et de voir quels effets

pour reconstituer le parcours de l’un des terroristes du Bataclan dans le métro et extraire les images afin de répondre à la réquisition judiciaire. Nous avons apporté des garanties en commission, en particulier en rendant ce dispositif expérimental et en limitant son champ à l’extraction et à l’exportation des données, si bien que ces logiciels ne sauraient, d’eux mêmes, assurer une sélection d’images ; celle ci relève d’un acte d’enquête.

peut paraître anodine, plus l’analyse de l’image est sophistiquée et même automatisée, plus on bascule dans l’acte d’enquête, qui est une prérogative exclusive des officiers de police judiciaire. Autre exemple, la duplication du cadre prévu dans la loi sur les jeux Olympiques semble disproportionnée pour ce qui concerne la vie de tous les jours. Enfin, une autorisation du préfet n’est pas envisageable dans la mesure où il s’agit, pour la RATP et la SNCF,

vérifications et des identifications concernant des demandeurs et des détenteurs de visa. Les agents de la Suge et du GPSR n’ayant aucune prérogative leur permettant de contrôler l’identité des voyageurs, et encore moins de vérifier la régularité du séjour sur le territoire de ceux ci,

Depuis l’intégration dans le droit français des dispositions issues de la réglementation européenne sur la protection des données personnelles, les services de sécurité de la RATP et de la SNCF ne sont plus autorisés à procéder à la collecte et au traitement de données sensibles. Cependant, ces informations sont nécessaires dans le cadre de communications réalisées tant au sein de ces services internes qu’avec les services de police et de gendarmerie. Le traitement de certaines de ces données sensibles permet d’identifier plus efficacement des individus présumés auteurs d’infractions, ce qui limite le risque d’erreur et évite potentiellement des actes de récidive.

en cas d’infractions flagrantes. Or, tout comme la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l’intérieur, la commission des lois a constaté que l’article 31 de la loi Informatique et libertés prévoyait déjà, au bénéfice de toute personne morale ou physique et pour les seules infractions flagrantes, la faculté de traiter des données sensibles pour le compte de l’État, par dérogation au principe général d’interdiction de collecte et de traitement de telles données applicable aux personnes morales et physiques, en application de l’article 6 de la loi précitée et de l’article 9 du règlement général sur la protection des données En outre, considérant qu’aucune règle spécifique en matière de traitement des données sensibles ne trouve à s’appliquer aux services internes de la SNCF et de la RATP que de surcroît, aucune règle en vigueur ne leur interdit de le faire pour cette finalité, il n’apparaît pas opportun de prévoir un tel régime. Il serait d’autant plus dangereux d’admettre un tel régime particulier pour ces services de sécurité cela conduirait à la création d’une nouvelle dérogation attachée non plus à la finalité recherchée, mais à la nature du bénéficiaire, modifiant ainsi profondément les équilibres du RGPD comme de la loi dite Informatique et libertés. Au surplus, une telle évolution impliquerait, par ricochet, la nécessité de modifier les dérogations à l’interdiction du traitement de données sensibles pour chacun

permettant d’infirmer un tel constat et d’identifier un obstacle juridique à la collecte de données sensibles en cas de poursuite d’une infraction flagrante par ces agents Enfin, la rédaction proposée paraît inaboutie en ce qu’elle prévoit, en son dernier alinéa, la collecte de données sensibles pour le traitement d’infractions flagrantes, mais dans le cadre de la mission de prévention des agents de la Suge et du GPSR

En effet, à l’occasion d’actes délictueux, les victimes et témoins fournissent des éléments de description des auteurs des méfaits, qui peuvent comprendre diverses données dites sensibles. Or, avec l’intégration du RGPD dans le droit français, les services internes de sécurité ne peuvent plus les transmettre. Ainsi, les chances de retrouver l’auteur du fait délictueux et criminel sont grandement diminuées par le manque de données descriptives. En temps réel, l’individu en question peut encore se trouver sur le secteur de commission des faits et être repéré soit grâce à la vidéosurveillance, soit par les effectifs présents sur le terrain, qui peuvent patrouiller dans le secteur. Sans information sur les descriptifs physiques des personnes recherchées,

dans certains véhicules, notamment les autobus, pour les conducteurs. En cas de danger, ces derniers peuvent actionner une pédale permettant au centre de supervision d’écouter ce qui se passe dans l’habitacle.

En premier lieu, cet article contrevient au principe de proportionnalité des peines en matière pénale, qui prévoit que le législateur doit fixer une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’auteur. l’occurrence, le fait de mendier, d’uriner ou de cracher dans des espaces non réservés à cet effet est puni des mêmes peines que le fait de porter une arme à feu ou de refuser d’obtempérer…

Aussi le Conseil constitutionnel se réserve t il le droit, au titre du principe de proportionnalité des peines, de censurer « les dispositions législatives prévoyant des peines manifestement disproportionnées par rapport aux faits reprochés.

sur les quais et de cracher par terre. Tout est mélangé, rien n’est toléré. Permettez moi de vous le rappeler, mes chers collègues, les mendiants dits d’habitude étaient punis de trois mois d’emprisonnement dans le code pénal de 1810.

Outre la prévention des troubles à l’ordre public, elle permet l’amélioration de l’attractivité des réseaux de transport et, par conséquent, favorise le report modal nécessaire à la transition écologique.

ont pu être recensés en 2023, contre 96 083 en 2015. S’il serait disproportionné de délictualiser une simple infraction aux règlements de la police du transport, la répétition à de multiples reprises d’une même infraction,

les usagers, les faire figurer dans le droit pénal semble un trop grand pas. Au delà de la problématique de l’intentionnalité de ces nouveaux délits, qui n’est pas résolue dans la rédaction

de 3 750 euros. La commission est attachée à préserver le caractère fortement dissuasif du délit d’incivilité d’habitude. En l’occurrence, l’effet dissuasif serait très diminué, voire annulé,

Certes, punir la répétition de ces comportements d’une peine de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende peut paraître sévère. Pour autant, les dispositions de cet amendement contiennent un effet de bord. auraient pour effet d’abaisser la répression actuellement prévue par le code des transports en cas de voyage habituel sans titre de transport valable. Or ce délit ne soulève pas de difficultés particulières et il n’existe aucune raison de le modifier. Pour cette raison, j’émets un avis défavorable

précise du champ de l’infraction, elle est de nature à assurer le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la sanction, ainsi que la proportionnalité de la peine. Nous avons déjà franchi un pas important avec la création de ce délit d’incivilité d’habitude, puisque, auparavant, la récidive de ces infractions contraventionnelles n’était pas sanctionnée en tant que telle. D’ailleurs, la fongibilité des infractions n’existe pas dans le régime contraventionnel existant : avoir reçu une amende pour une infraction aux règles de la police du transport n’aggrave pas la sanction encourue en cas de commission d’une autre infraction. aggravation pour le délit que nous créons, nous mettrions en place une disposition totalement inédite dans notre droit pénal et à la constitutionnalité mal assurée.

Je fais appel à votre expertise d’usage, car vous prenez peut être comme moi le TGV pour rejoindre vos circonscriptions. Fumer sur les quais de la gare est un usage que je constate chaque semaine. Chaque semaine, dès que le TGV qui me ramène à Montpellier s’arrête à la gare de Valence ou de Nîmes, des voyageurs, mais aussi des contrôleurs de la SNCF, en profitent pour descendre fumer une cigarette. Lorsque je me rends à la gare de Lyon, les mêmes agents de la SNCF et des entreprises auxquelles certains marchés ont été confiés, mais également les agents de la Suge, sont les premiers à « griller une cigarette » avec les voyageurs.

la mendicité restait prohibée dans les cours ou bâtiments de gares en vertu de l’article 85 du décret n° 42 730 du 22 mars 1942. Le décret du 3 mai 2016, relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics, précise dans le même sens que « la mendicité est interdite sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains » – article 11, alinéa 3. L’article 20 dudit texte précisait que le fait de pratiquer la mendicité sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la

De nombreuses associations, telles la Ligue des droits de l’Homme et la Fondation Abbé Pierre, attaquent régulièrement les arrêtés dits anti mendicité, le plus souvent de manière victorieuse.

puissance mondiale, aurait tout à fait les moyens d’éradiquer la misère. Mais que fait elle ? Elle répond à la mendicité par la répression : c’est un dramatique aveu d’échec ! Ni la mendicité ni la solidarité ne peuvent être considérées comme une infraction, et encore moins comme un délit. Où en sommes nous quand nos insuffisances en matière de solidarité nous poussent à cacher la misère en la refoulant de tous les espaces publics, notamment du train et des transports en commun ? Cet alinéa est particulièrement honteux.

si ! Vous oubliez de préciser que la mendicité sur le domaine public ferroviaire et routier est interdite et punie aujourd’hui d’une contravention de quatrième classe, respectivement au titre des articles R. 2241 16 et R. 3116 8 du code des transports. Nous souhaitons

M. Philippe Tabarot. Le présent amendement vise à élargir la liste des délits pouvant donner lieu à une peine complémentaire portant interdiction de paraître dans les réseaux de transport aux délits commis en matière de police ferroviaire. L’objectif est de prononcer cette peine à l’encontre des personnes ayant, par exemple, cherché à faire dérailler des véhicules ou à provoquer leur collision. Il semble en effet préférable d’interdire à des individus ayant commis de tels délits l’accès à certains réseaux, afin de garantir la sécurité de tous.

Ne pensez vous pas que le contrevenant sera d’autant moins incité à se faire connaître rapidement et à éviter ainsi l’immobilisation dans tout le périmètre de sécurité

Il convient de rappeler que les infractions d’imprudence ou de négligence, c’est à dire non intentionnelles, constituent l’exception dans notre droit répressif, et sont en principe réservées aux situations les plus graves – décès ou blessures importantes, par exemple. Je suis donc favorable à ces

permet déjà de réprimer ces faits en infligeant aux cas extrêmes cette sanction. J’ai vérifié. C’est d’ailleurs ce que la SNCF signale sur les titres. Si l’alerte n’a pas eu de conséquences sur le trafic, l’oubli relève de l’indemnité forfaitaire, soit quelques centaines d’euros.

? Cet amendement a pour objet d’accorder aux entreprises de transport public un accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. L’administration a déjà accès à ce fichier pour contrôler la moralité des personnes en contact avec les mineurs. Le Gouvernement comprend l’intention des auteurs de cet amendement. Toutefois, sa rédaction ne convient pas, dès lors que les entreprises de transport ne prennent pas de décisions administratives. Cet amendement pourrait donc être retravaillé dans le cadre de la navette.

des modalités de sélection des personnes morales de droit privé, qui seraient amenées à récolter des données fiscales et sociales sensibles auprès des administrations publiques et des organismes de sécurité sociale dans les cas de recouvrement des sommes dues pour les contraventions. les agents chargés du recouvrement habilités à communiquer des données fiscales et sociales doivent être des agents assermentés des opérateurs de transport, dûment formés en matière de protection des données à caractère personnel.

ne permet pas de connaître précisément les personnes qui pourront être désignées comme compétentes pour procéder à la saisie de ces données à caractère personnel ni de connaître avec précision les modalités de contrôle de l’administration. En l’absence de ces garanties, que, par exemple, la police, la gendarmerie ou les douanes sont en train de mettre en place – à l’inverse de nous –, il est préférable que la loi fixe directement les conditions et les modalités des contrôles opérés. La commission considère que cet amendement n’est pas opérant, dans la mesure où ce décret est prévu par l’article L. 2241 2 1 du code des transports, dans sa version en vigueur.

et de la RATP nous semble juridiquement fragile. Je rappelle que les emprises de transport restent des lieux publics. Veillons, là encore, à respecter les équilibres du continuum de sécurité. Je rappelle également que le droit prévoit un certain nombre d’outils, comme, pour les contrôleurs et les agents de sûreté, la possibilité de relever l’identité des contrevenants distinguer du contrôle d’identité –, ainsi que la possibilité, si ces derniers refusent, d’en aviser sans délai un OPJ et de les obliger à demeurer à disposition le temps nécessaire à l’information et à la décision de celui ci, en application de l’article L. 2241 2 du code des transports.

attestant son identité, afin que puisse être vérifiée la concordance entre celle ci et l’identité mentionnée sur son titre de transport. L’article 19 doit, enfin, permettre aux contrôleurs et aux agents de sûreté de vérifier l’exactitude des adresses relevées auprès de l’administration fiscale.

la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, dont les avis sont toujours particulièrement avisés. Je vous demande, mes chers collègues, de voter cette proposition de loi, parce qu’elle est attendue par les acteurs de terrain, par ceux qui sont en première ligne et – on l’a souvent dit – qui risquent leur vie au quotidien pour essayer d’améliorer la qualité des services de transport en général. J’ai une pensée également pour tous les usagers qui galèrent au quotidien et qui nous demandent d’améliorer l’offre ferroviaire. Or améliorer l’offre ferroviaire, c’est améliorer la qualité du service. Celle ci passe par

et de combler les lacunes de la législation pénale en vigueur. Cela dit, il est difficile à notre groupe de négliger l’équilibre entre la sécurité et les libertés publiques. Certains dispositifs nous ont alertés, ainsi que Véronique Guillotin l’a souligné lors de la discussion générale. Nous avons salué les travaux de la commission, qui avaient gommé une partie des défauts sécuritaires du texte initial, notamment en supprimant les articles 10 et 11. L’article 1 avait également été réécrit, sur l’initiative de notre rapporteure, dans une rédaction acceptable et mesurée. En revenant en partie à la rédaction initiale du texte, notre assemblée a donc pris la décision de rompre l’équilibre qu’elle avait su pourtant créer. Bien entendu, nous continuons de considérer qu’une partie des dispositions que nous avons votées ce soir sont nécessaires

prévention, dissuasion et répression ». Du fait qu’il s’agit d’une proposition de loi, les articles du texte ne tiennent pas cet équilibre. Quelques uns de ces articles reprennent des dispositions de sécurité globale qui ont été soumises à des réserves d’interprétation par le Conseil constitutionnel.

Merci